Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

Il est donc nécessaire de transformer en profondeur notre modèle agricole ; il est important que nous apportions collectivement des réponses à ces questions et à ces enjeux.